en application de l'article 5 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, qu'il lui confère, pour une durée de six mois, les prérogatives attribuées aux commissions d'enquête pour mener une mission d'information sur le contrôle des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Il a été donné connaissance de cette demande au Sénat lors de la séance du 8 février dernier. Je mets aux voix la demande de la commission des affaires sociales. la demande de la commission des affaires sociales. En conséquence, la commission des affaires sociales se voit conférer, pour une durée de six mois, les prérogatives attribuées aux commissions d'enquête pour mener cette mission d'information. Le Gouvernement sera informé de la décision qui vient d'être prise par le Sénat. L'ordre du jour appelle la discussion en deuxième lecture du projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, ratifiant les ordonnances prises sur le fondement de l'article 13 de la loi n° 2019-816 du 2 août 2019 relative aux compétences de la Collectivité européenne d'Alsace

Merci nous sommes réunis ici ce matin pour examiner ce projet de loi inscrit dans le prolongement de la loi du 3 août 2019 qui a, vous le savez, acté la création de la Collectivité européenne d'Alsace (CEA). Avec l'adoption de cette loi « Alsace », le Gouvernement a su créer un cadre de confiance pour mener à bien cette cette réforme importante et répondre à des besoins largement exprimés par les Alsaciens et les élus locaux. La loi du 3 août 2019 est le fruit de la volonté de l'État de reconnaître la particularité de ce territoire alsacien, territoire français profondément européen.

pour l'exercice de ses responsabilités dans des domaines aussi stratégiques que la gestion des infrastructures et le transport routier. Les ordonnances dont le Gouvernement vous propose la ratification sont le résultat de longs mois d'échanges et d'une concertation étroite avec les acteurs locaux, que je tiens à remercier.

CEA prévoyait l'adoption d'ordonnances. Il s'agit, d'abord, de donner la possibilité à la CEA de mettre en place une taxe sur le transport routier de marchandises sur certaines voies de son domaine public routier. Les Alsaciennes et les Alsaciens attendent, vous le savez, cette mesure depuis plus de quinze ans. L'article 1 du projet de loi que vous allez examiner procède à la ratification

Il s'agit, enfin, de préciser les conditions dans lesquelles la Collectivité européenne d'Alsace ou l'Eurométropole de Strasbourg continuent d'assurer les engagements de l'État portant sur les routes qui leur sont transférées et qui sont liées à la mise en service de l'autoroute A355. C'est chose faite avec l'article 3.

Avec ce projet de loi de ratification, le Gouvernement se fixe un cadre juridique clair tout en laissant d'importantes marges de manoeuvre à la CEA, par exemple sur la fixation des paramètres de la taxe sur le transport routier. Il s'agit de permettre l'adaptation des cadres aux contextes locaux.

La mise en oeuvre de la contribution au niveau de la CEA, potentiellement au 1 janvier 2024, préfigurera les travaux pour les autres collectivités volontaires, qui feront l'objet d'un processus. J'entends que les processus peuvent sembler longs.

que l'examen parlementaire de ce texte aboutisse dans le calendrier que vous connaissez. Mesdames, messieurs les sénateurs, l'adoption de ce texte est pleinement nécessaire à l'effectivité des ordonnances prises en 2021. Il s'agit d'un projet de longue date qui a fait l'objet d'un dialogue réunissant État et élus locaux dans un travail de concertation étroit,

Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, le texte sur lequel nous avons à nous prononcer aujourd'hui en deuxième lecture s'inscrit dans une démarche de long terme engagée par les Alsaciennes et les Alsaciens voilà plus de quinze ans. Ce texte comptait initialement trois articles visant à ratifier trois ordonnances, dont l'une a plus particulièrement fait l'objet de débats nourris en première lecture : l'ordonnance à l'instauration d'une taxe sur le transport routier de marchandises par la Collectivité européenne d'Alsace. Depuis 2005 en effet, date de la mise en place d'une taxe sur le transport de marchandises en Allemagne, l'Alsace souffre d'importants reports de trafic sur le réseau routier qui la traverse. Ces reports sont source d'importantes nuisances environnementales et affectent aussi la santé des riverains. Après de multiples tentatives législatives pour instaurer une taxe sur le transport de marchandises français, dont nous n'avons oublié les rebondissements, l'une des trois ordonnances que le présent projet de loi vise à ratifier porte notamment sur la possibilité donnée à la Collectivité européenne d'Alsace de mettre en place une telle taxe sur le domaine routier qui lui a été transféré. En première lecture, en commission puis en séance publique, le Sénat avait considérablement enrichi le dispositif prévu par l'ordonnance, en introduisant une vingtaine d'articles additionnels sur ce sujet, suivant trois axes. Premier axe, nous avions cherché à renforcer l'efficacité et le caractère opérationnel du dispositif prévu dans l'ordonnance du 26 mai 2021, afin notamment de le rendre facilement transposable à d'autres collectivités.

Le deuxième axe de progrès proposé par le Sénat pour améliorer ce texte portait sur les conditions d'un meilleur dialogue entre les collectivités territoriales directement ou indirectement concernées.

Nous avons donc veillé à favoriser, en amont de sa mise en place, la création d'une instance de concertation entre les collectivités et, en aval, une évaluation des reports de trafic. Troisième et dernier axe : nous avions, en première lecture, veillé à anticiper la révision de la directive Eurovignette dans un double objectif : d'une part, faire en sorte que la taxe puisse prendre en compte les émissions de CO2 des véhicules, afin d'améliorer sa dimension environnementale et, d'autre part, permettre à la Collectivité européenne d'Alsace, d'appliquer la taxe aux véhicules utilitaires légers à partir de 2,5 tonnes. Nous avions bien évidemment prévu que ces évolutions soient mises en oeuvre sous réserve de l'entrée en vigueur de la nouvelle version de la directive Eurovignette. Au terme de son examen en première lecture au Sénat, le texte comptait ainsi 23 nouveaux articles, en plus des trois articles du projet de loi initial. Ces évolutions résultent d'un important travail d'écoute et de concertation, y compris au plus près du terrain, en Alsace. Après son examen à l'Assemblée nationale, le texte nous revient avec 21 articles, dont deux nouveaux articles introduits sur l'initiative de l'Assemblée nationale. En définitive, il apparaît que l'Assemblée nationale a globalement conforté les apports du Sénat puisqu'elle en a conservé une grande partie. Dix des articles additionnels créés au Sénat ont été adoptés conformes ou modifiés à la marge à l'Assemblée nationale. Ainsi, ont été conservés les articles relatifs à la création d'un comité de concertation des collectivités territoriales en matière de taxation des poids lourds, ou encore l'aggravation des sanctions en cas de comportements frauduleux. D'autres articles introduits par le Sénat ont fait l'objet de modifications plus importantes, mais qui ne remettent pas en cause leurs objectifs, comme l'article 1, qui permet à la Collectivité européenne d'Alsace de mettre en place une solution de pour les redevables occasionnels de la taxe. J'ai également dialogué avec mon collègue rapporteur à l'Assemblée nationale pour définir des positions de compromis sur quelques dispositions. S'agissant de l'évaluation de la taxe, par exemple, nous avions souhaité prévoir la remise d'un rapport d'étape après deux ans de mise en oeuvre. L'Assemblée nationale a supprimé ce rapport d'étape, mais, faisant preuve d'un esprit de compromis, a en contrepartie réduit de cinq ans à trois ans le délai accordé au Gouvernement pour remettre un rapport d'évaluation au Parlement. Les députés ont également enrichi le texte de deux nouvelles dispositions qui permettent encore, à la marge, d'améliorer le caractère opérationnel de l'ordonnance. Je viens d'évoquer des points positifs, dont on peut se réjouir. Ceux-ci ne doivent néanmoins pas occulter un certain nombre de reculs sur des apports du Sénat, qui se traduisent par la suppression de six articles insérés au Sénat et la modification de plusieurs autres. Par exemple, les articles adoptés au Sénat afin d'anticiper la révision de la directive Eurovignette ont été supprimés, l'Assemblée estimant qu'ils portaient atteinte à la lisibilité du droit. Je ne souscris pas à cet argument, et je rappelle que l'entrée en vigueur des dispositions en question était subordonnée à la révision de la directive. Je regrette ces censures qui constituent des reculs significatifs sur certains apports du Sénat. Je vous propose néanmoins, mes chers collègues, d'adopter ce texte conforme à celui qu'a adopté l'Assemblée nationale en première lecture, pour trois raisons principales. D'abord, comme je vous l'ai indiqué, je constate que le travail du Sénat n'a pas été dénaturé, ses principaux apports ayant été conservés par l'Assemblée nationale. Ces apports permettent sans aucun doute d'améliorer significativement les ordonnances, et donc de renforcer le caractère opérationnel d'un dispositif attendu depuis longtemps par les Alsaciens. Je vous propose donc, par l'adoption d'un texte conforme, d'accompagner la Collectivité européenne d'Alsace dans sa démarche. Dans l'absolu, il serait certes envisageable de faire évoluer ce texte afin de rétablir certains articles, mais j'en viens justement à mon deuxième point : le calendrier parlementaire rend difficile d'envisager une troisième lecture, compte tenu de la suspension à compter du 28 février prochain. Par

au milieu du gué, et avec pour conséquence le fait que l'ordonnance, déjà entrée en vigueur, ne serait ni modifiée ni ratifiée. Très concrètement, si nous n'adoptions pas ce texte conforme, la Collectivité européenne d'Alsace serait privée de la possibilité de mettre en place une solution de paiement pour les redevables occasionnels. Mais non ! pour le comité de concertation préalable ou encore le rapport évaluant les potentiels reports de trafic. Cette option est peu opportune, car elle conduirait à ne retenir aucun des apports du Sénat, qui ont pourtant fait l'objet d'un important travail de concertation. Soit, et c'est l'option pour laquelle je plaide aujourd'hui, nous choisissons d'adopter ce texte conforme à celui adopté par l'Assemblée nationale afin de préserver les apports des deux chambres qui permettent, comme je l'ai évoqué, de renforcer le caractère opérationnel du dispositif et de créer les conditions du dialogue entre les collectivités territoriales. Enfin, troisième point, l'adoption d'un texte dans les mêmes termes que celui adopté par l'Assemblée nationale permettra de ratifier les trois ordonnances du projet de loi, et donc de sécuriser leurs dispositions en leur conférant une valeur législative. La taxe alsacienne est susceptible de faire l'objet de plusieurs contentieux. Une sécurisation de l'ordonnance par sa ratification est donc opportune pour renforcer ce dispositif. Pour l'ensemble de ces raisons, je vous propose, mes chers collègues, dans un esprit de responsabilité, d'adopter ce texte sans modification. La parole

Pour le Parlement européen, ce sera peut-être le moment du vote définitif de la refonte de la directive relative aux redevances routières, autrement dit la directive Eurovignette, transformée par le compromis du 15 juin dernier, insatisfaisant de mon point de vue, qui encadre les conditions dans lesquelles les États peuvent instaurer Pour notre Sénat, c'est donc à présent la deuxième lecture de la loi ratifiant l'ordonnance pour la mise en place de la taxe poids lourds en Alsace. Cette taxe alsacienne devrait être, en dehors des autoroutes concédées à péage, le seul périmètre où s'appliquerait dans notre pays un dispositif relevant de cette directive. Sauf si, à partir de 2024, des régions frontalières décidaient d'utiliser la possibilité de taxer les poids lourds que leur a ouverte la loi Climat et résilience. Autrement dit, dans une perspective européenne d'harmonisation et de renforcement du principe pollueur-utilisateur-payeur pour le fret routier, c'est l'Alsace qui sera, selon la façon de voir les choses, soit l'exception durable, comme un petit village gaulois atypique qui aurait enfin la capacité de résister à l'afflux de nuisances camionnées, soit la pionnière d'une extension, voire d'une généralisation, à venir. Que l'un ou l'autre scénario l'emporte, la mise en oeuvre alsacienne doit être de toute façon facilitée et accompagnée. Elle a besoin de l'action efficace de l'État pour franchir sans tarder les obstacles et les étapes qui sont encore devant elle avant qu'une taxe à la hauteur de la allemande ne la protège effectivement, comme elle le veut depuis dix-sept ans. Pour la protéger, ce qui doit être fait est clair : une taxe alsacienne d'un niveau équivalent à celui de la taxe allemande. Rappelons-le, l'Allemagne, comme la Suisse qui a été pionnière en la matière, n'a pas détruit avec sa taxe les équilibres économiques de ses entreprises de transport. Elle a, au contraire, modernisé sa logistique, amélioré sa performance économique, optimisé ses charges transportées, abondé les moyens d'un report modal qui permet un fret ferroviaire allemand quatre fois plus important que le nôtre et mis en place une stratégie de transition des transports que nous lui envions. Je parlais à l'instant de la nécessité d'une action efficace de l'État ; je dois donc relever, madame la secrétaire d'État, que si ces ordonnances avaient été publiées par le Gouvernement dans les délais prévus par la loi « Alsace nous ne serions pas contraints aujourd'hui à un vote conforme obligatoire en deuxième lecture pour tenir le calendrier parlementaire qui s'achève la semaine prochaine. C'est dommage, car s'il faut saluer le travail des rapporteurs du Sénat et de l'Assemblée, des améliorations étaient, à mon avis, encore à notre portée, pour mieux s'adapter aux possibilités de la directive nouvelle, comme cela a été dit. Je pense à la lutte contre l'abus des véhicules utilitaires légers assurant du transport pour le compte d'autrui, ou encore à la meilleure prise en compte des riverains du sillon lorrain. C'est dommage. Les conditions précipitées et contraintes de ce travail parlementaire risquent paradoxalement d'aboutir ce matin à empêcher une belle unanimité- il y aura peut-être une petite part de votes négatifs, ce qui est regrettable -sur cette avancée positive concernant une Alsace pleinement volontaire et tellement impatiente.

Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, il s'agit ici non pas de refaire le débat que nous avons eu en première lecture, mais de porter une appréciation sur le travail d'adaptation conduit par notre rapporteur. Les adaptations proposées nous semblent conformes aux Je tiens à mon tour à saluer la qualité du travail produit sous l'égide de notre collègue Jean-Claude Anglars. C'est aussi la raison pour laquelle nous n'avons déposé aucun amendement. Pour autant, cela ne modifie en rien l'appréciation que nous portons au fond sur ce texte et sur la régionalisation de l'écotaxe, qui ne nous paraît pas être la bonne réponse à un problème pourtant bien réel. Nous comprenons l'impatience des collectivités d'Alsace et, au-delà,

de recueillir quelques subsides pour compenser ces effets et de pouvoir contribuer au développement de modes de transport alternatifs à la route. Pour autant, la régionalisation de l'écotaxe ne nous paraît pas être la bonne solution, car toutes les régions de France ne sont pas géographiquement égales.

nous considérons que la réponse au problème rencontré passe aussi par la mobilisation de moyens importants pour développer le fret ferroviaire. En effet, le mode ferroviaire, qui est écologiquement le plus vertueux, est le seul mode de transport qui paye la totalité de ses coûts

j'ai envie de dire : enfin ! Effectivement, au regard des spécificités du trafic routier en Alsace, caractérisé par un report important de flux de circulation de poids lourds en provenance d'Allemagne à la suite de la mise en place d'une- la fameuse taxation des poids lourds -sur l'autoroute allemande, le transfert décidé en 2019, et effectif depuis le 1 janvier 2021, de la voirie nationale non concédée à la CEA offre la perspective d'une gestion homogène du trafic et de ses contraintes. L'enjeu qui nous réunit aujourd'hui est de pourvoir la collectivité des outils nécessaires à l'exercice de cette nouvelle compétence de façon pragmatique. Je dirais même que, fort opportunément, tous les paramètres convergent donc avec la loi Climat et résilience d'août 2021 qui permet la mise en place d'écotaxes régionales dans les territoires subissant des reports significatifs de circulation d'agir concrètement sur le flux de transport routier de marchandises et, par voie de conséquence, de peser positivement sur la transition écologique. En effet, l'Alsace subit depuis de trop nombreuses années une dégradation importante de ses infrastructures routières, assortie d'une paralysie du trafic à certaines heures. Il en découle une accidentologie élevée, même parler des effets délétères pour la santé publique dus à la forte augmentation de la pollution de l'air et du bruit. Aussi, en tant que sénateur du Bas-Rhin, et me faisant la voix du territoire que je représente, je me réjouis d'assister

Nous ne pouvons donc que nous inscrire dans la ligne constructive qui a prévalu tout au long du processus d'adoption de ce projet de loi. À ce titre, je salue tout particulièrement, avec les égards qu'il mérite, le rapporteur Jean-Claude Anglars pour son investissement et ses travaux de qualité. Certes, tout n'est pas parfait et quelques ajustements pratiques n'ont pas permis d'atteindre un consensus total. que la CEA ne puisse pas installer un dispositif de contrôle automatisé, ce qui est regrettable. Mais retarder l'adoption d'un texte tant attendu sur le territoire aurait constitué un manquement particulièrement préjudiciable, d'autant que, globalement, ce texte qui arrive au terme de son processus législatif accorde à la CEA une grande souplesse pour adapter ses outils à la réalité de terrain. Je me réjouis donc de l'occasion qui nous est offerte aujourd'hui et apporte donc bien évidemment mon entier soutien au projet de loi de ratification, qui représente un premier test.

Je ne minimise pas pour autant certaines problématiques qui ne vont pas manquer d'alimenter durablement les débats. Je pense notamment aux transporteurs locaux français qui vont être fortement pénalisés, mais également aux reports vers des axes secondaires gratuits qui vont naturellement et inexorablement avoir lieu. Mais j'ai confiance dans le dialogue qui va s'instaurer pour dégager des solutions permettant de traiter de manière pragmatique et différenciée l'ensemble de ces situations-

votera donc aujourd'hui la ratification de ces ordonnances, qui représentent une avancée importante pour l'Alsace tout en répondant aux préoccupations de nos citoyens en matière de changement climatique. La parole

organisée par la Communauté européenne d'Alsace portant sur la question de son maintien au sein de la région Grand Est. Voilà les effets d'un découpage régional dont personne ne voulait. C'est sûr ! Oui à la différenciation, non aux entorses à l'indivisibilité de la République et à l'égalité de nos concitoyens devant la loi Des garde-fous identiques doivent être instaurés pour tous les territoires. Le groupe du RDSE, qui avait d'ailleurs voté contre la création de la CEA, fait siennes les craintes exprimées dans les départements limitrophes quant à la mise en place de la taxe poids lourds, dont les modalités d'application sont définies par le présent projet de loi, largement amélioré par le Sénat. Le territoire de la CEA n'est pas le périmètre le plus pertinent pour la mise en oeuvre de cette taxe qui, à défaut d'être instituée au niveau national afin de permettre un financement territorialement équitable de l'ensemble des infrastructures de transport, devrait être instaurée au niveau régional, comme le permettra ultérieurement l'article 137 de la loi Climat et résilience votée en juillet dernier. Ce texte ouvre la voie à un pouvoir fiscal des collectivités territoriales à géométrie variable, ce que nous ne pouvons pas approuver. Nous comprenons l'impatience de nos collègues alsaciens.

engendrant des nuisances pour les habitants dont la qualité de vie est fortement affectée. Néanmoins, nous considérons que la taxe ne fera que déplacer le problème tant que les autres territoires ne pourront pas s'en saisir.

demandait l'application concomitante de la taxe sur cet axe. Bravo ! Les émissions de gaz à effet de serre ne baisseront donc pas si l'on n'accélère pas la décarbonation du secteur des transports.

je me réjouis particulièrement de la recommandation visant à affecter ces recettes aux investissements nécessaires à la transition écologique. En effet, cette transition ne peut pas reposer uniquement sur la fiscalité. D'autres solutions doivent être créées en parallèle, afin de n'entraver ni la compétitivité de nos entreprises ni le pouvoir d'achat des ménages. Le choix de l'écologie ne doit pas toujours être celui de la taxation ou de la punition ; une telle politique serait vouée à l'échec. Le financement de la politique du fret ferroviaire demeure très en retard. Des trains circulent sur des voies datant, à certains endroits, du XIX siècle. Si la taxe poids lourds est appliquée, encore faut-il qu'elle produise suffisamment de ressources pour financer le fret ferroviaire et mettre fin à la distorsion de concurrence qui bénéficie encore au transport routier. En France, le prix par kilomètre est 30 % plus cher que celui qui est appliqué en Allemagne. Réjouissons-nous de la fin du feuilleton législatif de la taxation des poids lourds, du moins pour le seul épisode alsacien.

l'application, enfin, pour la première fois en France, du principe « pollueur-payeur », dans ce drame français de l'écotaxe, parsemé de « bonnets rouges », de « gilets jaunes » et de sécessionnistes alsaciens. lieu au moment même où le Parlement européen votera la révision de la directive Eurovignette relative à la taxation des poids lourds pour certaines infrastructures.

ces mesures a été jonché de nombreuses embûches, de promesses gouvernementales sans cesse reniées et de trahison. Pour parvenir à leurs fins, des véhicules législatifs singuliers sont empruntés, comme le texte qui a porté sur les fonts baptismaux la Collectivité européenne d'Alsace, nouveau nom d'un grand et beau département possédant bien peu de compétences particulières véritable de ce texte est plutôt d'être le ferment de la division de la région Grand Est, sous un prétexte de différenciation. En témoignent les propos clivants et fracassants du Premier ministre à Strasbourg en janvier 2021,

il vous aurait été loisible de mépriser notre démarche en rendant ces amendements irrecevables. Vous ne l'avez pas fait, et je vous en remercie encore. Mais là,

avec la majorité gouvernementale, et en opposition avec la majorité régionale, qui pourtant demande ce texte ! Le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain votera contre.

il aura fallu prendre son mal en patience, mais après des années de transactions, d'avancées puis de renoncements, de valses-hésitations, nous sommes en train de franchir un pas décisif.

les logiques partisanes. Nous connaissons tous la situation : les autoroutes alsaciennes sont surchargées et dangereuses. Ce constat ne date pas d'hier, et la situation empire de jour en jour

En conséquence de cette saturation, les accidents ne cessent de faire l'actualité régionale. Pour ne prendre qu'un exemple récent, le 24 janvier dernier, à la suite d'un carambolage impliquant plusieurs véhicules au niveau de Sausheim dans le Haut-Rhin, l'A35 a été coupée pendant près de cinq heures. L'article 1 de ce projet va mettre fin à tout cela. Issu de l'article 13 de la loi relative aux compétences de la Collectivité européenne d'Alsace, le dispositif va permettre d'instaurer une taxe sur le transport routier de marchandises, et ainsi de désengorger cet axe autoroutier pris d'assaut par les poids lourds en transit, afin d'éviter la fameuse fameuse d'outre-Rhin. Toutefois, il va falloir faire montre d'encore un peu de patience : la décongestion de notre principal axe autoroutier ne devrait pas avoir lieu avant la fin de 2024. Pourquoi encore de longs mois d'attente ? Parce qu'il reste beaucoup de travail. Types de véhicules concernés, systèmes de contrôle choisis, acceptabilité auprès des transporteurs locaux, délai minimal des autorisations nécessaires : toutes ces modalités ne sont pas encore arrêtées.

en grand transit. Ces modalités techniques prennent du temps. Il s'agit d'un point important que la CEA doit prendre à bras-le-corps, mais le Parlement, et en particulier le Sénat, a souhaité les garantir, du moins pour partie. est l'objet des vingt-trois articles introduits au Sénat, qui ont été pour la plupart conservés par nos collègues députés. Je mentionnerai la possibilité pour la Collectivité européenne d'Alsace de moduler le taux kilométrique de la taxe en fonction des saisons, l'augmentation du montant des amendes infligées visant à éluder le paiement de la taxe ou de l'équipement électronique embarqué, l'inclusion des sociétés donneuses d'ordre dans la consultation préalable à l'instauration de la taxe, la création d'un comité pour faciliter la concertation des collectivités territoriales en matière de taxation des poids lourds. En revanche, nos collègues de l'Assemblée nationale ont procédé à quelques rectifications. Je pense notamment à la suppression de l'article instaurant l'écotaxe pour les grands véhicules utilitaires légers, qui pourrait ne pas correspondre à la réforme de la directive Eurovignette, ce qui n'est pas souhaitable, en matière de lisibilité et de droit. Par ailleurs, une telle disposition pénaliserait les entreprises locales qui disposent fréquemment de ce type de véhicules. Hormis quelques modifications, l'Assemblée nationale a largement repris les apports bénéfiques de notre Haute Assemblée, ce dont nous nous réjouissons. Pour conclure, mes chers collègues, il faut désormais aller vite ; pour cette raison, le vote conforme proposé nous convient. Il est urgent que la CEA s'empare rapidement des compétences accordées par la loi, pour définitivement mettre un terme aux caravanes de camions qui perturbent la vie de beaucoup de nos concitoyens alsaciens. La parole

Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, une fois de plus, le Parlement a démontré l'importance de la ratification des ordonnances. Très bien ! D'une part, l'Assemblée nationale et le Sénat ont pour prérogative majeure de contribuer à la fabrication de la loi. D'autre part, les améliorations apportées à ce projet de loi sont notables. Je salue ici l'important travail effectué par la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, et en particulier par son rapporteur. Je me réjouis que les avancées réalisées au Sénat aient été pour la plupart conservées lors de la première lecture à l'Assemblée nationale. Il est essentiel de maintenir certaines précisions quant à l'encadrement des mécanismes prévus par les ordonnances, à l'image des dispositions venant soit compléter les mécanismes de sanction et de constatation d'irrégularités dans le cadre de l'écotaxe, soit préciser les montants des amendes.

celui des effets de l'écotaxe sur les territoires limitrophes. Le rapport prendra en compte l'évaluation des reports de trafic sur le réseau du domaine public des régions, des départements et des communes limitrophes.

Nous serons amenés, quoi qu'il en soit, à nous emparer du sujet prochainement, une transposition de cette directive étant nécessaire. Cependant, nous pouvons d'ores et déjà nous réjouir que ce sujet soit abordé au niveau européen. Si ce projet de loi, que nous examinons pour la deuxième fois, n'est pas parfait, il comporte des avancées notoires. Nous garderons un oeil sur l'application de l'écotaxe et des divers mécanismes prévus, ainsi que sur leurs effets potentiellement négatifs. Nous sommes en présence d'un texte équilibré, et nous entendons les arguments du rapporteur demandant une adoption conforme. L'urgence de la situation et la demande du territoire nous conduisent, tout en restant vigilants, à être pragmatiques. Le groupe Les Indépendants votera en faveur de ce texte,

Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, nous nous retrouvons ce matin pour voter en deuxième lecture le projet de loi ratifiant les ordonnances relatives aux compétences de la Collectivité européenne d'Alsace. Je tiens tout d'abord à remercier M. le rapporteur Jean-Claude Anglars de son travail, ainsi que de son écoute attentive des élus locaux dans la préparation de ce texte. Je suis évidemment très favorable à la ratification de ces ordonnances, dont les mesures sont attendues depuis fort longtemps par les Alsaciens. Ce texte est important pour trois raisons : premièrement, il répond à des enjeux importants pour l'Alsace ; deuxièmement, il répond à une forte attente et à un engagement de longue date enfin, il répond au besoin de prendre en compte des spécificités locales et d'avancer dans la voie de la différenciation. Il s'agit de mettre en oeuvre les dispositions de la loi de 2019

celui de l'encombrement du sillon rhénan depuis la mise en place d'une taxe poids lourds sur l'A5 allemande au 1 janvier 2005. Depuis ce jour, des camions venus de toute l'Europe circulent sur l'autoroute A35, de Mulhouse à Strasbourg en passant par Colmar. Il s'agit donc de répondre à un besoin et à une réalité territoriale transfrontalière, car ce report engendre de nombreuses conséquences, comme la dégradation des infrastructures, une accidentologie élevée en raison du volume de circulation, mais également un fort impact environnemental. Vous le comprenez, mes chers collègues, il s'agit donc d'une réelle attente des élus alsaciens et de toute la population depuis plus de Ces ordonnances s'inscrivent également dans le cadre d'un engagement et d'une volonté politique ancienne, comme l'a rappelé notre collègue Claude Kern. Adrien Zeller avait déjà souhaité un tel dispositif pour l'Alsace. Puis, en 2005, c'est le député Yves Bur qui avait fait adopter par le Parlement une taxe sur le transit des poids lourds en Alsace, mais ce projet n'avait malheureusement pas été appliqué, et avait été abandonné en 2013. Aujourd'hui, nous y sommes enfin. Je me réjouis Je me réjouis que les apports du Sénat aient été conservés dans ce texte, notamment en ce qui concerne la création d'un comité de concertation des collectivités territoriales en matière de taxation des poids lourds, également au sujet du système de, solution technologique mise à la disposition de la collectivité pour la constatation et le paiement de la taxe, notamment pour les redevables occasionnels. occasionnels. Malgré l'abandon de certains apports significatifs, comme l'anticipation de la révision de la directive Eurovignette ou encore la possibilité pour la Collectivité européenne d'Alsace d'installer des dispositifs de contrôle automatisés, ce texte

d'un moment important, car ce texte concerne l'instauration de la taxe poids lourds tant espérée par une grande partie des Alsaciens. En effet, depuis 2006, nous attendons une amélioration de la circulation sur nos routes, pour plus de sécurité, moins d'embouteillages et une diminution des nuisances liées au trafic, comme le bruit et la pollution. d'un moment important pour les élus locaux, notamment pour les maires des communes concernées et pour les conseillers de la Collectivité européenne d'Alsace, qui ont fait avancer ce dossier. Cette taxe permettra une régulation optimale par la CEA

qui a provoqué un report du trafic des poids lourds en transit sur l'A35. Nous pouvons donc être satisfaits du texte examiné aujourd'hui, que l'Assemblée nationale a adopté à l'unanimité le 26 janvier dernier. Il s'agit là d'un texte de compromis, qui n'appelle pas de modifications. Ce texte de loi permettra à la Collectivité européenne d'Alsace, tout en respectant le cadre européen, d'être dotée de marges de manoeuvre sur les modalités de cette taxe, afin notamment de l'adapter aux spécificités de notre territoire. En effet, nous déterminerons alors notamment le tonnage minimal et les catégories de véhicules taxables, le réseau concerné, le taux kilométrique de la taxe en fonction des saisons, la majoration pour les coûts externes, ainsi que les réductions et les exonérations. Je tiens à préciser que la volonté de la CEA n'est pas de percevoir une quelconque recette fiscale supplémentaire. Il s'agit bien de mettre en place une gestion raisonnée du flux du trafic routier de marchandises sur certaines voies du domaine de la CEA, et de financer la dégradation des voiries causées causées par les véhicules lourds en transit, selon une logique d'utilisateur-payeur. Nous sommes également satisfaits de la conservation du en faveur des usagers occasionnels et de la souplesse du dispositif qui permet de ne pas pénaliser les transports régionaux. Des semaines de débats parlementaires ont permis d'améliorer les ordonnances, tout en respectant leur état d'esprit, c'est-à-dire le droit à la différenciation et les accords de Matignon. Il faut maintenant laisser le texte se déployer et faire ses preuves. Il servira de terrain d'expérimentation pour les autres régions de France. La CEA est prête à lancer les appels à projets,

Je salue, en tant que conseillère d'Alsace, le vote des députés qui ont donné leur feu vert à la mise en place de cette taxe poids lourd pour le transport routier de marchandises, communément appelée « écotaxe alsacienne », en ne modifiant qu'à la marge le texte que le Sénat avait adopté et enrichi en première lecture. Je ne reviendrai pas sur les péripéties de l'écotaxe en France, que tout le monde connaît, mais je me réjouis que nous puissions donner aujourd'hui à la Collectivité européenne d'Alsace la possibilité d'expérimenter une solution nouvelle en votant conforme, je l'espère, ce projet de loi.

à une attente et à une demande forte des Alsaciens, qui subissent au quotidien les nuisances liées au trafic des poids lourds. Il est cohérent de doter la CEA des moyens nécessaires à la mise en oeuvre d'une compétence qui lui est dévolue par la loi de 2019.

J'aimerais conclure sur une note positive : non seulement cette taxe répond aux enjeux sanitaires et écologiques, puisqu'elle désengorgera l'A35 et limitera la pollution atmosphérique, mais elle ouvre également la porte à la mise en place future d'autres dispositifs similaires dans d'autres territoires. Il s'agit d'une expérimentation inédite, qui mérite pour cette raison d'être soutenue. Nous devrions tous en espérer la réussite. Vous l'aurez compris, j'espère sincèrement que le Sénat votera conforme ce projet de loi. La discussion

transposition de la directive européenne concernant un fléau des transports qui n'est pas pris en compte par le texte actuel, lié aux véhicules utilitaires légers

entre conducteurs de VUL et conducteurs de poids lourd, pour ce qui concerne les temps de repos, ont été sensiblement atténués par l'adoption du paquet mobilité 1, qui limitera clairement les distorsions de concurrence dont pouvaient bénéficier ces VUL.

introduite. Toutefois, au fur et à mesure de nos échanges avec le rapporteur de l'Assemblée nationale, nous sommes parvenus à une position d'équilibre concernant la question du bilan de la taxe. Si l'Assemblée nationale avait initialement simplement supprimé le rapport d'étape adopté par le Sénat, elle a ensuite, en contrepartie de cette suppression, réduit le délai de remise d'un rapport du Gouvernement au Parlement de cinq ans

taxe kilométrique sur les véhicules de transport routier de marchandises sur le seul territoire alsacien aura pour principale conséquence le report d'une partie du trafic sur l'autoroute lorraine A 31, même si mes collègues alsaciens ne veulent pas le reconnaître.

Même si la loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets permet au Gouvernement, d'ici deux ans, de légiférer par ordonnance pour permettre aux régions de mettre en place des contributions spécifiques sur le transport routier de marchandises, il faut agir sans attendre pour permettre, dans l'intervalle, à la région Grand Est

lequel prévoit la remise au Parlement d'un rapport présentant le bilan de la mesure en matière de maîtrise du trafic routier de marchandises. Il s'agit d'intégrer la problématique de l'A31 aux conclusions de ce rapport. À cet égard, je veux remercier ma collègue alsacienne

quatre raisons principales. Premièrement, la loi Climat et résilience prévoit déjà la possibilité pour les régions volontaires de mettre en place cette taxe ... Dans deux ans ! Il appartiendra donc aux régions volontaires et, on l'espère, à la région Grand Est de s'en saisir, une fois que les routes leur auront été transférées, si elles le souhaitent. Deuxièmement, il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Il semble en effet important que la région, comme l'a fait la CEA, prenne le temps d'élaborer son propre dispositif, en coconstruction avec les services de l'État. Une telle démarche doit s'inscrire dans un calendrier défini, pour en garantir le succès. Troisièmement, ces amendements ne respectent pas l'article 34 de la Constitution. En effet, il n'est pas constitutionnel de fixer par décret le régime et les conditions de l'application d'une taxe. Un certain nombre de modalités relèvent du domaine de la loi : l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement.

Vous le savez, le président de la CEA, la Collectivité européenne d'Alsace, a décidé de recourir à l'association de la population pour la mise en oeuvre de ses politiques, quelles qu'elles soient. S'est d'ailleurs terminée la nuit dernière une votation

toutes les étapes de préparation, auxquelles il a été fait allusion, de mise en place des décisions précisant les tonnages, les catégories, le réseau taxable exact, les dispositifs kilométriques, les majorations pour coûts externes, les possibilités de la directive Eurovignette, les réductions et les exonérations. Toutes ces étapes devront se réaliser au mieux, pour tenir la promesse d'une entrée en vigueur sans perte de temps, dans un délai raisonnablement réduit, et garantir- c'est très important -le caractère transférable d'un dispositif, qui, comme me le disait hier M. le ministre chargé des transports, doit être un modèle pionnier.

du présent texte. J'informe le Sénat que la commission mixte paritaire chargée d'élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi visant à renforcer le contrôle parental sur les moyens d'accès à internet est parvenue à l'adoption d'un texte commun. L'ordre du jour appelle la discussion en nouvelle lecture de la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, visant à combattre le harcèlement scolaire

Monsieur le président, monsieur le vice-président de la commission, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, cette proposition de loi est le dernier texte sur l'éducation de la législature. Aussi, permettez-moi de remercier les représentants de la Nation que vous êtes pour leur travail continu et leur engagement sincère sur les sujets d'éducation. Je me réjouis aussi que ce soit précisément cette proposition de loi visant à combattre le harcèlement scolaire que nous ayons à examiner aujourd'hui, d'abord parce que la lutte contre le harcèlement en milieu scolaire aura été l'une des grandes causes de mon action pendant ce quinquennat, ensuite parce qu'il s'agit d'un sujet qui, comme souvent lorsqu'il est question de l'école, a vocation à créer de la concorde et à nous rassembler.

Nous l'avons accueillie favorablement, comme nous l'avons fait chaque fois que des propositions allaient dans le bon sens- et ce fut souvent le cas, je tiens à le souligner, de la part des représentants de la chambre haute. La lutte contre le harcèlement, nous en sommes tous d'accord, est un enjeu de société. Cet enjeu dépasse largement le cadre scolaire et nécessite une mobilisation générale ; il renvoie tout simplement à la valeur de fraternité qui est le ciment de notre nation. Si les actions menées depuis 2017 ont permis de contenir le harcèlement « physique » entre élèves, la progression rapide et exponentielle du cyberharcèlement nous appelle à redoubler d'efforts et de vigilance. Nous ne nous habituerons jamais à ce que des vies d'enfants et d'adolescents soient brisées, abîmées, parfois de façon irrémédiable, par ce fléau. Nous lutterons donc sans relâche et avec la dernière énergie contre ce phénomène. En la matière, nous avons d'ailleurs beaucoup avancé. Nous ne nous résignerons pas. Nous pouvons atteindre un objectif de zéro harcèlement à l'école, c'est possible ! Certains pays, certains établissements, certains professeurs y réussissent chaque jour, y compris en France. Cet objectif est donc à notre portée. Et je me réjouis que cette proposition de loi nous permette d'avancer en ce sens. Du plan de lutte contre le harcèlement à l'école, en 2018, à la généralisation du programme de lutte contre le harcèlement à l'école (pHARe), en 2022, nous n'avons pas attendu pour prendre à bras-le-corps ce phénomène. Dès 2018, nous avons engagé un plan volontariste et ambitieux pour combattre le harcèlement à l'école autour de trois grands axes

le dialogue avec les plateformes de réseaux sociaux, le lancement de cinq campagnes de prévention autour des thèmes suivants :, rôle des témoins, dynamiques de groupe, école primaire, cyberharcèlement.

C'est pourquoi le ministère finance deux numéros d'écoute, le 3020 pour le harcèlement et le 3018 pour le cyberharcèlement, en partenariat avec l'association e-Enfance.

C'est pourquoi nous avons travaillé à améliorer la prise en charge des situations de harcèlement en renforçant la formation initiale et continue des professeurs, qui intègre désormais cette dimension de façon systématique, et en développant le dispositif des élèves ambassadeurs, qui permet la

programme pHARe à toutes les écoles et à tous les collèges. Celui-ci s'inspire en partie du programme finlandais KiVa, la Finlande faisant partie des pays qui ont particulièrement bien réussi dans le domaine de la lutte contre le harcèlement. Notre pays peut devenir ainsi un exemple de ce qui se fait de mieux au monde en la matière. Très concrètement, nous dotons les établissements d'un référent harcèlement, de personnels formés à la détection et au traitement des situations, ainsi que d'élèves ambassadeurs pour le signalement. Ce programme est déjà une réalité sur le terrain, dans une bonne partie des établissements. Les familles sont associées à cet effort collectif, la mise à disposition de ressources accessibles en ligne

La méthode utilisée, appelée Pikas, a fait ses preuves, car elle permet aux adultes de repérer les « signaux faibles » et d'intervenir rapidement pour protéger les victimes, tout en amenant les auteurs à une prise de conscience. Lorsque vient le moment de la sanction, en effet, il est souvent déjà trop tard ... Une méthode s'applique, donc, établissement par établissement, avec des équipes formées et un traitement de chaque situation. L'objectif est très simple : aucun cas de harcèlement ne doit rester sans réponse. Si nous voulons lutter efficacement contre le harcèlement en milieu scolaire, nous devons sortir d'une logique exclusivement défensive pour passer à l'offensive, ce qui revient à dire que nous menons une politique du « climat scolaire En effet, le harcèlement est d'une certaine façon le résultat d'une dégradation du climat scolaire. Ce que nous devons viser, c'est tout simplement l'installation d'un climat scolaire fraternel, à base d'engagement notamment. Avec le Conseil d'évaluation de l'école, que nous avons créé par la loi pour une école de la confiance, nous sommes désormais en mesure d'évaluer le climat scolaire dans chaque établissement, afin de disposer d'un état des lieux et, le cas échéant, de prendre des mesures adéquates. Il nous faut également chercher à promouvoir l'engagement des élèves, leur sens de l'intérêt général, du civisme et de l'empathie, ces « compétences douces » qui sont si importantes.

cela va de pair avec le renforcement de l'enseignement moral et civique et de l'éducation aux médias et à l'information. Nous avons par ailleurs créé, outre les ambassadeurs « Non au harcèlement », 250 000 écodélégués, afin de diversifier les formes d'engagement des élèves.

en bout de chaîne, le service national universel (SNU) et les services civiques, à 16 ans et au-delà, qui constituent une forme d'accomplissement du parcours citoyen, avec un effet rétroactif sur tout ce qui précède- le service national universel, rappelons-le, permet d'envoyer un signal quant à l'engagement des élèves en amont du SNU lui-même. C'est la raison pour laquelle j'ai souhaité que de jeunes engagés en service civique puissent être mobilisés pour participer à la mise en oeuvre du programme pHARe dans les écoles et les établissements- ce sont souvent ces jeunes qui parlent le mieux aux élèves de tels sujets. sujets. La proposition de loi qui vous est soumise vient donc couronner cette dynamique générale. Elle apporte une nouvelle pierre à l'édifice, en élargissant la base légale du harcèlement scolaire, que nous avions déjà commencé à poser la loi pour une école de la confiance, et en créant un délit spécifique de harcèlement scolaire. Sur plusieurs autres points, elle complète l'action engagée à travers le programme pHARe notamment. Je pense en particulier au rôle des associations, dont certaines ont participé activement à l'élaboration de ce dispositif. Elle permet surtout, mesdames, messieurs les sénateurs, d'envoyer un message très clair à la Nation tout entière : non, le harcèlement n'a pas sa place dans nos établissements. Oui, l'école doit rester, selon la fameuse formule de Jean Zay, cet « asile inviolable où les querelles des hommes

création d'une fonction de directeur d'école- là aussi, le Sénat a pris toute sa part ... La liberté et l'égalité ont donc été des clés de notre politique scolaire. Avec cette proposition de loi, on voit aussi que la troisième valeur de notre devise républicaine est au centre de l'action menée. Cette valeur si

manqué voilà quinze jours ! -, mes chers collègues, à l'occasion de cet examen en nouvelle lecture de la proposition de loi visant à combattre le harcèlement scolaire, permettez-moi de vous faire part, au nom de la commission, de satisfactions et de regrets. Je commencerai par les points de satisfaction. Le texte élaboré en première lecture par la Haute Assemblée est le fruit d'un travail consensuel. Il a rassemblé opposition et majorité sénatoriale autour d'un objectif commun : agir globalement pour lutter contre le harcèlement scolaire.

J'ai tenu, lors de l'élaboration du texte en première lecture, à m'appuyer le plus possible sur ces travaux et à reprendre les recommandations à portée législative du rapport. Ainsi de la prise en compte des témoins, du renforcement de la formation initiale et continue de l'ensemble des adultes d'un établissement, des actions résolues contre le cyberharcèlement ou encore de l'instauration d'une sensibilisation annuelle des élèves. Ces travaux ont permis également d'éclairer nos débats sur l'opportunité de créer un délit spécifique de harcèlement scolaire. Ce consensus transpartisan s'est également traduit dans les amendements que nous avons adoptés. Ils émanent de plusieurs groupes politiques, et notamment de l'opposition sénatoriale. En voici quelques exemples

demandé permettra notamment de dresser le bilan du « chèque psy » destiné aux mineurs et aux étudiants, annoncé par le Président de la République dans le cadre du confinement. Autres exemples : une prise en compte de la lutte contre le harcèlement scolaire par le réseau des établissements français à l'étranger, l'étranger, l'obligation pour les réseaux sociaux de mieux sensibiliser leurs utilisateurs contre le cyberharcèlement. Des amendements de la majorité sénatoriale ont été soutenus par l'opposition.

Le Sénat avait proposé des assouplissements de la carte scolaire, ainsi que des modalités de recours à l'instruction en famille, pour les élèves victimes de harcèlement. Un élève harcelé qui quitte son établissement, c'est toujours une défaite de l'école, je l'ai dit et redit. Mais, dans certains cas, la poursuite de la scolarité dans l'établissement où il a été harcelé pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, n'est pas possible ou pas souhaitée par la victime. Certes, la loi confortant le respect des principes de la République prévoit la possibilité de commencer rapidement l'instruction en famille d'un enfant victime de harcèlement scolaire, sans attendre l'autorisation de l'administration, qui peut prendre deux mois. Mais cette situation demeure transitoire.

L'ensemble de ces éléments démontre une volonté commune des membres de la Haute Assemblée de voter un texte ambitieux, permettant une lutte globale contre le harcèlement scolaire et le cyberharcèlement. J'ai donc d'autant plus de regrets quant à l'échec de la commission mixte paritaire. Deux points durs opposent le Sénat et l'Assemblée nationale : l'extension de la définition du harcèlement scolaire aux fins d'y inclure des faits commis par des adultes ; la création d'un délit spécifique de harcèlement scolaire. Pourquoi ces deux dispositions nous posent-elles problème ? J'y reviendrai plus en détail à l'occasion de la présentation de la question préalable déposée par la commission. Voici néanmoins quelques éléments, afin de faire taire les rumeurs selon lesquelles le Sénat se serait opposé à un texte de lutte contre le harcèlement scolaire. L'élargissement de la définition du harcèlement scolaire, monsieur le ministre, risque d'affaiblir l'institution scolaire, dans un contexte de défiance envers l'école. Le droit existant permet déjà de sanctionner pénalement et administrativement des actes de harcèlement commis par des adultes sur les élèves. Quant au délit spécifique, son quantum de peine semble disproportionné et en définitive peu opérant. Quelle est la signification de peines si élevées, qui ne seront sans doute pas appliquées dans les faits ? Nous étions prêts à un compromis sur l'un de ces points. Malheureusement, nos collègues députés n'étaient pas disposés à faire un pas vers nous pour que nous les retrouvions au milieu du gué. Le texte a été examiné en nouvelle lecture le 10 février dernier à l'Assemblée nationale. Que reste-t-il de nos apports ? Trop peu de choses peu de choses ! L'Assemblée nationale a bien entendu rétabli sa définition du harcèlement scolaire, ainsi que la création d'un délit pénal spécifique. Elle acte ses positions, qui divergent des nôtres, sur ces deux points essentiels pour le Sénat.

envoyons clairement un message de lutte contre ce fléau qui amplifie le harcèlement scolaire et ne laisse à la victime ni répit ni abri, pas même dans la sphère privée. Par ailleurs, l'Assemblée nationale a refusé toute possibilité d'assouplissement des modalités de dérogation à la carte scolaire ou de recours à l'instruction en famille pour l'élève harcelé. Elle a supprimé de la liste des personnes bénéficiant d'une formation initiale et continue à la prévention et à la lutte contre le harcèlement scolaire les titulaires d'un contrat d'engagement éducatif.

Faute de financement pérenne, cette nouvelle mission risque de se transformer très rapidement en nouvelle charge financière. Espérons que des crédits budgétaires soient prévus dans le prochain budget afin de reconduire les 1 600 référents sur lesquels l'Assemblée compte pour la mise en oeuvre de cette nouvelle mesure.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, en première lecture, j'avais déjà souligné le caractère plus symbolique qu'opérant de cette proposition de loi.

que l'existence des réseaux sociaux et des plateformes aggrave, mérite clairement que l'on fasse mieux. Le calendrier imposé n'est pas non plus propice à un examen serein de cette proposition de loi et il est regrettable que l'ensemble, ou presque, des dispositions adoptées par le Sénat aient été balayées.

nous interpelle. On ne saurait mettre sur un pied d'égalité des harceleurs mineurs et des adultes responsables détenteurs d'une autorité et soumis par ailleurs à un cadre statutaire strict. est des Crous, on impose à un opérateur en difficulté budgétaire, dont les référents harcèlement ne seront plus financés à partir de septembre prochain, de remplir une mission que leur ministère de tutelle ne semble pas avoir songé à leur confier

quitte, comme l'écrivait Colette Mélot dans son rapport, à « nuire à la nécessaire mobilisation générale ». Nous ne comprenons pas la volonté des députés d'adopter un quantum de peine qui risque de n'être jamais appliqué tant il est disproportionné par rapport au droit commun. il faut mieux, beaucoup mieux lutter contre le harcèlement qui intervient dans le cadre scolaire en renforçant les instruments juridiques existant dans notre droit, en cohérence avec celui-ci. De ce point de vue, faire du harcèlement scolaire une circonstance aggravante du harcèlement nous semble particulièrement sensé. Comme cela a été souligné, l'efficacité de la lutte contre le harcèlement scolaire passe par l'action systémique et conjuguée des différents acteurs de la communauté éducative. À ce propos, il manque dans cette proposition de loi des éléments centraux de la mobilisation contre le harcèlement : des moyens pour la médecine scolaire, l'amélioration de la prise en charge psychologique et psychique des élèves, la mise en sécurité d'urgence des élèves harcelés.

un tiers seulement des enseignants se sentent suffisamment armés pour cela et 83 % d'entre eux indiquent n'avoir jamais reçu aucune formation ni information sur la détection du harcèlement scolaire et l'accompagnement des victimes. Quant aux multiples enjeux qui doivent être abordés en éducation morale et civique- environnement, laïcité, lutte contre le harcèlement, et j'en passe -, leur énumération suffit à démontrer qu'il est impossible

les dispositions de cette proposition de loi viennent en percuter les objectifs, sans rien améliorer. Il est donc regrettable que nos deux chambres n'aient pas trouvé de terrain de conciliation sur ce sujet qui mérite pourtant notre pleine et entière mobilisation,

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle lecture de la proposition de loi visant à combattre le harcèlement scolaire. Je souhaite exprimer ma déception quant à l'échec de la commission mixte paritaire sur un sujet qui s'annonçait pourtant transpartisan et ne prête guère à polémique. Pour mémoire, le harcèlement scolaire et le cyberharcèlement concernent entre 800 000 et 1 million d'enfants ; en d'autres termes, 6 % à 12 % des élèves subissent ou ont subi une forme de harcèlement au cours de leur scolarité. Chacun d'entre nous doit prendre conscience de cette réalité et mesurer le drame, individuel et collectif, que le harcèlement représente aujourd'hui pour l'école de la République. Nous parlons d'enfants ou d'adolescents durablement affectés par les menaces, les humiliations ou les violences physiques dont ils font l'objet. Le texte qui nous vient de l'Assemblée nationale comporte à nos yeux plusieurs écueils. Le premier concerne le cyberharcèlement. Lors de l'examen du texte en première lecture au Sénat, nous nous étions attachés à y intégrer ce phénomène trop absent de la version issue des travaux de l'Assemblée nationale. Le cyberharcèlement crée un continuum du harcèlement scolaire, les réseaux sociaux, les tablettes ou les smartphones, ne laissant aucun répit aux victimes. Il amplifie également l'aspect « meute » du phénomène. Je rappelle que, selon les chiffres de la mission d'information sénatoriale sur le harcèlement scolaire et le cyberharcèlement, près d'un quart des collégiens y sont confrontés.

Le second point concerne la définition du harcèlement scolaire introduite par l'Assemblée nationale, qui a souhaité ne pas limiter le harcèlement scolaire à un harcèlement entre pairs. Cette définition, incluant les adultes, est un très mauvais signal envoyé aux personnels de l'éducation nationale. Elle va à rebours des textes que nous avons défendus dans cet hémicycle- je pense par exemple à la proposition de loi créant la fonction de directeur d'école. Cette définition ne fera que renforcer un climat de défiance de plus en plus insupportable pour les personnels de l'éducation nationale et déconstruire un peu plus l'autorité des professeurs. Un autre point de désaccord majeur concerne la création d'un délit spécifique dans le code pénal. Nous ne sommes pas convaincus de la portée pédagogique de ce dispositif, qu'invoquent les députés, et craignons plutôt qu'il n'engendre une incohérence dans les peines applicables, voire une rupture d'égalité. Comme l'avait dit ma collègue Annick Billon lors de l'examen du texte en première lecture, ne laissons pas croire que la création d'un nouveau délit suffira à résoudre le problème. Si tel était le cas, nous aurions déjà pu le régler sur la base des textes existants. Enfin, en supprimant du texte les articles 3 A, 3 B et 3 C, l'Assemblée nationale refuse toute possibilité d'assouplissement des dérogations à la carte scolaire, disposition défendue par nombre de nos collègues.

Nous regrettons que les recommandations de cette mission d'information n'aient pas été prises en compte dans l'élaboration du texte que nous examinons aujourd'hui. Mes chers collègues, vous l'aurez compris, le groupe Union Centriste, dans sa très grande majorité, votera la motion tendant

Ce fléau continue de se répandre, malheureusement aidé par les outils numériques, le cyberharcèlement en étant l'une des formes les plus violentes. Il est favorisé par le silence des victimes, motivé souvent par la peur ou la honte et par le silence des témoins. C'est pourquoi je me réjouis du choix de l'Assemblée nationale de conserver un apport du Sénat : l'intégration des témoins, aux côtés des victimes et des auteurs de harcèlement, dans les mesures prises par les établissements, afin de lutter contre le harcèlement scolaire. Les députés ont également décidé d'inclure une formation à l'identification et à la prise en charge des témoins dans la formation initiale à destination des adultes à même d'être confrontés à des faits de harcèlement scolaire : personnels médicaux et paramédicaux, personnels de l'éducation nationale, travailleurs sociaux et animateurs, mais aussi policiers, gendarmes et magistrats. Car, on le sait, le témoin est un personnage central du phénomène de harcèlement. Il s'agit d'un phénomène de groupe, et le harceleur trouve parfois son intérêt à harceler dans la présence de témoins, auditoire de l'humiliation qu'il fait subir. Nous devons encourager cette démarche d'implication du témoin pour qu'à l'avenir il ne soit plus simplement passif, mais qu'il devienne un allié dans le combat mené contre ce mal meurtrier qu'est le harcèlement scolaire. La définition même du harcèlement scolaire dans le code de l'éducation a été l'un des principaux points de désaccord. Je ne crois pas qu'il faille exclure les adultes du champ du harcèlement scolaire. L'article 1 de la proposition de loi consacre le droit à une scolarité ou à une formation sans harcèlement. C'est une affirmation qui se veut de portée générale, protégeant l'ensemble des élèves et des étudiants à l'égard de leurs pairs, mais aussi à l'égard de toutes les personnes travaillant au sein de l'établissement d'enseignement. Exclure une catégorie de personnes enverrait un message confus et affaiblirait la portée de cette affirmation. Cette limitation a pu être motivée par une volonté de protéger les enseignants d'éventuels recours abusifs de la part d'élèves et de leurs familles. Au contraire, c'est bien un moyen de protéger les enseignants que de renvoyer les plaignants devant la justice, qui constituera un recours protecteur. Le second élément de désaccord a été la création d'un délit autonome de harcèlement scolaire. Créer un délit spécifique, inscrit dans le code pénal, est un signal fort à destination des auteurs de harcèlement scolaire. Il peut déclencher une prise de conscience de la gravité des actes commis, surtout chez de jeunes auteurs. Aussi, il est logique que le quantum de peine proposé ouvre la possibilité de poursuivre tout auteur de harcèlement scolaire sur une base unique, qui prend en compte la réalité des conséquences du harcèlement scolaire et sa gravité.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je veux vous dire ici ma forte déception face à l'absence d'accord en commission mixte paritaire sur cette proposition de loi visant à combattre le harcèlement scolaire, dont j'ai salué le dépôt en première lecture et que nous n'avons eu de cesse d'améliorer durant la navette. La responsabilité en incombe principalement à l'Assemblée nationale et à sa majorité, qui n'a absolument pas souhaité avancer vers des solutions de compromis. Cette attitude est à l'image de celle du Gouvernement, qui a, hélas ! fait peu de cas du rapport de la mission d'information sénatoriale sur le harcèlement scolaire et le cyberharcèlement, que j'ai eu l'honneur de présider, et dont la rapporteure était Colette Mélot.

Le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain a accueilli plutôt favorablement cette proposition de loi en première lecture, principalement comme outil de mobilisation de l'ensemble de la société face à ce fléau, sans ignorer cependant la portée purement symbolique de certaines dispositions de ce texte. Le nerf de la guerre contre le harcèlement scolaire, ce sont les moyens octroyés à l'éducation nationale pour recruter davantage de médecins, d'infirmières, de psychologues scolaires. Je regrette l'insuffisance de ces moyens, monsieur le ministre, alors que ces acteurs sont en première ligne pour lutter contre le fléau du harcèlement scolaire, comme j'ai eu l'occasion de vous le dire lors de la présentation du rapport de notre mission sénatoriale. Cette proposition de loi contient incontestablement des dispositions positives, comme la place donnée dans le code de l'éducation à la lutte contre le harcèlement scolaire, et l'extension de la définition du harcèlement scolaire au harcèlement universitaire. Positifs aussi l'application des nouvelles dispositions de lutte contre le harcèlement aux établissements privés, le renforcement de la formation et de la sensibilisation de l'ensemble des personnels au contact des élèves, ou encore la saisie du matériel ayant servi au harcèlement. Je regrette que l'Assemblée nationale n'ait pas accepté la réécriture de l'article 4 de ce texte, proposée par le Sénat sur l'initiative de la rapporteure pour avis de la commission des lois. En effet, nous ne sommes pas favorables à la création d'un délit spécifique de harcèlement scolaire, et nous trouvions que sa transformation en circonstance aggravante du délit de harcèlement était une bonne solution de compromis. Le délit spécifique de harcèlement scolaire tel que l'Assemblée nationale le propose est assorti de peines particulièrement lourdes et totalement inapplicables. Notre mission d'information sénatoriale avait d'ailleurs préféré miser sur une meilleure prévention. Autre regret, l'Assemblée nationale est revenue sur la rédaction de l'article 7 de la proposition de loi, en retirant l'ajout de notre groupe qui prévoyait un renforcement du concours des hébergeurs et fournisseurs d'accès à la lutte contre le harcèlement. Nous proposions la présentation périodique aux utilisateurs de vidéos de sensibilisation aux bons usages du numérique et à la prévention du cyberharcèlement, avec mention des peines encourues par les contrevenants et voies de recours pour les victimes, conformément aux préconisations de notre mission sénatoriale. Quelques avancées proposées par le Sénat ont été conservées par l'Assemblée nationale, comme la prise en charge des témoins de faits de harcèlement au même titre que les victimes ou les auteurs, ou encore l'affirmation du rôle central des visites médicales dans l'identification des enfants victimes. Je me félicite également de l'introduction au Sénat de dispositions permettant le recrutement des assistants d'éducation en après six ans d'activité, tout en regrettant que cette mesure de bon sens ne s'applique pas aux accompagnants d'élèves en situation de handicap (AESH). C'est une différence de traitement injuste, incompréhensible et génératrice d'une colère légitime de ces personnels ô combien indispensables ! Notre groupe n'était pas en accord avec la totalité de la version sénatoriale de la proposition de loi. Ainsi, nous n'étions pas favorables à l'ajout de dispositions concernant l'instruction en famille, le harcèlement scolaire pouvant servir de prétexte pour renforcer ce mode d'instruction que nous considérons comme inégalitaire. Nous désapprouvions aussi l'exclusion du champ du texte des faits de harcèlement en provenance des enseignants ou du personnel des établissements : c'est un phénomène certes minoritaire, mais qui doit être considéré. Nous saluons aussi le rétablissement de l'article 6, supprimé au Sénat, qui prévoit des stages de sensibilisation aux risques liés au harcèlement scolaire dans le cadre de stages de citoyenneté ou de formation civique, comme le souhaitait notre mission sénatoriale. Je suis sûre qu'il aurait été possible de conjuguer les apports positifs de l'Assemblée nationale et du Sénat sur ce texte, et je regrette que cela n'ait pas été possible, en grande partie- je le répète -du fait de l'attitude dogmatique de la majorité à l'Assemblée nationale. tendant à opposer la question préalable, car il est opposé par principe à l'arrêt des débats, en particulier sur ce sujet qui préoccupe fortement nos concitoyens et qui touche nos enfants. Il aurait préféré pouvoir débattre en détail des différents points que je viens d'évoquer et voter en faveur du texte élaboré par l'Assemblée nationale qui, malgré sa frilosité et son aspect abusivement répressif, constituait tout de même une avancée pour lutter contre le harcèlement scolaire et le cyberharcèlement. La parole est à Mme Nadège Havet.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, à la suite de l'échec de la commission mixte paritaire, nous examinons pour la dernière fois la proposition de loi de notre collègue député Erwan Balanant visant à combattre le harcèlement scolaire,

mieux protéger les enfants et les jeunes adultes tout au long de leur parcours éducatif, de la maternelle jusqu'à la vie universitaire. Autant d'avancées nécessaires face à l'ampleur du phénomène et à sa gravité, puisque certaines victimes vont parfois jusqu'à se donner la mort. sont en effet toujours trop nombreux à être victimes de tels actes et à en souffrir, dans l'enceinte de l'établissement et/ou sur les réseaux sociaux. Je tiens à saluer ici, une nouvelle fois, le travail de nos collègues Sabine Van Heghe et Colette Mélot

Il bride la liberté individuelle, porte atteinte à l'égalité en droits et fracasse l'idéal de fraternité. » Oui, chaque année, plus de 700 000 enfants sont cassés, abîmés par le harcèlement scolaire. C'est ce chiffre effroyable que rappelle sur son site l'association Les Papillons. Ces enfants peuvent être les nôtres, nos nièces, nos neveux, nos cousins, nos voisins. Nous sommes toutes et tous concernés et touchés. Je le disais en première lecture, qui d'entre nous regarderait son enfant se débattre dans ses cauchemars, dans ses peurs, perdre confiance en lui et dans les adultes ? Nous nous devons d'agir et beaucoup a été fait depuis 2017, comme vous l'avez rappelé, Dans la continuité de ces actions, notre groupe avait souhaité inscrire ce texte à son ordre du jour réservé. Nous avions déposé plusieurs amendements de rétablissement en première lecture, ici même en séance publique, car la version initiale du texte, votée de façon transpartisane par l'Assemblée nationale, nous semblait plus efficace. Parmi les dispositions adoptées en commission au Sénat, nous avions notamment regretté l'exclusion des adultes de la définition du harcèlement scolaire, et sa limitation aux pairs, de même que la suppression du délit autonome de harcèlement scolaire et sa transformation en circonstance aggravante. Nous sommes favorables à l'intégration d'une mention explicite, dans le code pénal, de la sanction du harcèlement scolaire et universitaire en tant que tel. Et nous sommes donc favorables à son rétablissement par l'Assemblée nationale. Nous partageons également pleinement le maintien à l'Assemblée nationale de l'article 3 , introduit cette fois au Sénat par Mme Toine Bourrat et plusieurs de nos collègues. Celui-ci vise à modifier l'article du code de l'éducation relatif aux conditions de recrutement et d'emploi des assistants d'éducation. Il prévoit ainsi la définition par décret des conditions dans lesquelles l'État peut conclure un contrat à durée indéterminée avec un assistant d'éducation (AED). C'est une avancée importante que nous approuvons. Enfin, nous ne voterons pas la motion tendant à opposer la question préalable, puisque nous n'en partageons pas l'objet, mais il est exact, au regard des conclusions de la commission mixte paritaire et de son déroulement, que de nouvelles avancées semblent compromises. La parole

et s'il est un lieu qui devrait être un sanctuaire pour nos enfants, c'est bien l'école, lieu de transmission des savoirs et de socialisation. Entre 800 000 et 1 million d'élèves sont victimes chaque année en France de harcèlement scolaire. Pour ces enfants, le havre se transforme en geôle et l'étau se resserre parfois jusqu'à la mort. En 2021, vingt-deux enfants sont décédés des suites de harcèlement. Agir contre la violence, c'est semer les graines d'une société de la bienveillance dans laquelle le respect de l'autre accompagne le respect de soi-même, comme vous l'avez souligné, monsieur le ministre. Cette proposition de loi est le fruit du travail mené par Erwan Balanant, dans le cadre de la mission gouvernementale qui lui a été confiée. En tant que rapporteure de la mission sénatoriale contre le harcèlement

qui prend le plus souvent naissance dans le harcèlement à l'école, en l'amplifiant, ait disparu du texte, alors que cette dimension dématérialisée prend une ampleur grandissante.

Si notre rapport n'a pas emprunté la voie de la réponse judiciaire, la demande de création d'un délit autonome de harcèlement scolaire vient d'une volonté des acteurs de terrain, confrontés chaque jour à cette violence insupportable. Nous pouvons le comprendre. Mon souhait est pourtant de favoriser autant que possible la prévention, la détection et le traitement des situations de harcèlement scolaire. Cette proposition de loi intègre une partie des propositions de la mission d'information sénatoriale : le stage de sensibilisation, la formation des professionnels et la mise à contribution des plateformes, notamment. L'État n'est pas seul à bord. L'ensemble de la société doit se mobiliser. Pour cela, je souhaite que le prochain gouvernement érige la lutte contre la violence à l'école en grande cause nationale. Nous devons agir plus particulièrement sur « le dernier kilomètre », en utilisant sur le terrain des dispositifs existants. Sensibiliser les élèves, les enseignants et les parents dès la rentrée scolaire me paraît primordial. La médecine scolaire a un rôle central à jouer dans la détection des situations de harcèlement. Or la pénurie de médecins qui touche de nombreux territoires entrave l'accès à la santé physique et psychologique de nombreux élèves. Nous devons aussi prendre en charge l'après-harcèlement, en favorisant le remboursement d'un panier de soins indispensables pour accompagner les élèves victimes. Des stages pour renforcer l'estime de soi et apprendre des techniques de négociation et de gestion des conflits pourraient être proposés à ces élèves. Nous devons progresser ensemble, en nous inspirant des initiatives vertueuses, aux échelles locale, nationale et européenne. Placer la parole et la confiance au centre des apprentissages, faire en sorte que le chemin de l'école soit celui du vivre ensemble, retrouver le sens de notre destin collectif, telle est la ligne d'horizon qui doit nous guider, avec une seule certitude : la honte doit changer de camp, pour que la jeunesse reste ce champ des possibles dans lequel chacun peut trouver sa place, grandir, étudier, s'épanouir dans le respect des valeurs qui fondent notre République. Ne nous trompons donc pas de cible en tombant dans un arbitrage politique ! En dépit des réserves qui sont les miennes

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, rapporteure pour avis lors de la première lecture de la proposition de loi qui nous réunit ce matin, j'ai pu auditionner les représentants d'associations de défense des victimes du harcèlement scolaire et je tiens à leur manifester tout mon soutien, tout comme je pense à ces jeunes adolescents victimes, harcelés par leurs pairs et qui vivent l'enfer. Rappelons que la mission d'information du Sénat sur le harcèlement scolaire et le cyberharcèlement, présidée par notre collègue Sabine Van Heghe et dont la rapporteure était Colette Mélot, avait souligné en septembre dernier la nécessité d'une prise de conscience et d'une action rapides face à l'ampleur de ce phénomène. Selon les chiffres donnés par cette mission, 6 % à 10 % des élèves subiraient une forme de harcèlement au cours de leur scolarité, et un quart des collégiens seraient confrontés à du cyberharcèlement. Au total, chaque année, entre 800 000 et 1 million d'enfants seraient victimes de harcèlement scolaire. Terrible constat ! Il est de notre devoir de lutter contre toutes les formes de harcèlement, et notamment le cyberharcèlement, qui prend une place de plus en plus importante dans notre société. Mais n'oublions pas que la priorité est d'éduquer ces jeunes afin qu'ils respectent leurs camarades, et d'aider à la libération de la parole afin que toute violence verbale, physique, psychologique ou numérique soit dénoncée. Pour ce faire, le rôle des parents est primordial. Je tiens à revenir sur le point majeur d'achoppement avec nos collègues de l'Assemblée nationale lors de la commission mixte paritaire, et plus particulièrement sur le titre II de la proposition de loi, dont la commission des lois s'était saisie. Tout en partageant, bien entendu, le souhait d'améliorer le droit pénal pour lutter contre le harcèlement scolaire, la commission a suivi les orientations de la mission d'information sénatoriale sur le harcèlement scolaire et le cyberharcèlement, et refusé l'inscription dans la loi d'un délit autonome de harcèlement scolaire. Nous ne négligeons pas l'enjeu symbolique, mais le champ de l'infraction spécifique et le quantum de peine proposé nous ont paru problématiques et surdimensionnés. Nous avons néanmoins reconnu l'importance de réprimer les faits de harcèlement qui interviennent dans les établissements d'enseignement, donc scolaires ou universitaires. Mais, en cohérence avec la position de la commission de la culture du Sénat et de son rapporteur, Olivier Paccaud, nous les avons limités aux faits de harcèlements entre pairs. Il est regrettable que les députés se soient opposés à la rédaction du Sénat concernant les personnes susceptibles de commettre l'infraction de harcèlement scolaire. Le Sénat refuse l'inclusion dans la définition du harcèlement scolaire des faits commis sur un enfant par un adulte, pour la simple et bonne raison qu'ils sont déjà inscrits dans la loi. Par ailleurs, l'extension aux adultes, prévue par l'article 1 initial de la proposition de loi, risquerait de provoquer une instrumentalisation du délit de harcèlement par des élèves ou des parents d'élèves en conflit avec l'enseignant, et de contribuer à l'affaiblissement de l'autorité de ce dernier. Lors de l'examen du projet de loi pour une école de la confiance, le Gouvernement et la commission avaient d'ailleurs été défavorables à l'inclusion dans la définition du harcèlement scolaire de faits commis par des adultes. Le Sénat, dans sa très grande majorité, a donc souhaité réintégrer le harcèlement dans les établissements d'enseignement comme une circonstance aggravante du délit général de harcèlement prévu par le droit existant. Même si notre objectif est le même et si les autres divergences qui existent sur le titre II ne sont pas essentielles, notre désaccord sur la question du délit spécifique est majeur. Nous regrettons que le Gouvernement et l'Assemblée nationale n'aient pas entendu, une nouvelle fois, la voix du bon sens. Est-il nécessaire de surlégiférer en permanence ? Pourquoi ne pas simplement compléter le droit existant ?

Je tiens à saluer le lancement, le 8 février dernier, de l'application 3018 visant à lutter contre le cyberharcèlement. C'est un premier pas, mais, dans le combat contre le cyberharcèlement, la France ne peut agir seule. L'Europe doit se saisir de ce sujet grave et inciter les plateformes à jouer leur rôle dans la lutte contre cette violence quotidienne et sournoise. Les plateformes ont le devoir de prévenir ces faits et d'augmenter leur réactivité pour retirer les contenus participant au cyberharcèlement La présidence française du Conseil de l'Union européenne pourrait être l'occasion de prendre ce sujet à bras-le-corps. Les voyages diplomatiques du Président sont nécessaires, mais trouver des solutions concrètes à ce problème de société me paraît également prioritaire. Profitons de ce semestre pour montrer l'exemple J'informe le Sénat que la commission mixte paritaire chargée d'élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi relative au choix du nom issu de la filiation n'est pas parvenue à l'adoption d'un texte commun.